que nous ont dit nos concitoyens à cette occasion ? Qu'ils voulaient plus de démocratie. Avec ce texte, monsieur le secrétaire d'État, votre réponse est : moins de démocratie sociale, moins d'instances représentatives avec moins de prérogatives et moins de représentants du personnel. Élu du département de la Loire, je pense forcément aujourd'hui à Jean Auroux : il avait créé les CHSCT, en 1982, pour favoriser le dialogue entre employeurs et employés sur la question fondamentale de la santé et des conditions de travail. Cette instance représentait aussi un progrès parce qu'elle mettait la prévention au coeur de ses travaux. Après quelque trente années de fonctionnement, cette institution est désormais l'une des plus dynamiques de notre pays. Les élus qui y siègent sont devenus très compétents sur des sujets extrêmement variés et complexes. Monsieur le secrétaire d'État, vous voulez vous passer de ces compétences au moment même où vous allez généraliser la précarité dans la fonction publique.

De même, l'insécurité et l'instabilité du travail augmentent la fréquence des risques psychosociaux chez les travailleurs précaires. Pour faire face à ces risques accrus, vous supprimez l'instance la plus adaptée, et vous la remplacez par une

Assassi, sur l'article. À l'heure où nous débattons des CHSCT, les anciens dirigeants de France Télécom sont entendus par la justice à la suite de suicides ou de tentatives de suicide, de dépressions et de burn-out du personnel causés par une restructuration mortifère. Quel est donc le signal envoyé par le Gouvernement aux directions de la fonction publique ? À l'instar de l'ordonnance relative au dialogue social du 22 septembre 2017, ce projet de loi porte atteinte à la représentation du personnel par la fusion des instances de représentation au sein des comités sociaux. Créé- je le rappelle à mon tour -par l'une des lois Auroux de 1982, le CHSCT constitue un véritable progrès social pour les travailleuses et les travailleurs ; et il n'a cessé de monter en puissance ces dernières décennies. On pense notamment au rôle essentiel que ces structures ont joué dans la lutte contre des projets de réorganisation néfastes pour la santé physique et mentale des personnels, et leurs conditions de travail, mais aussi à leur rôle de lanceur d'alerte pour protéger nos concitoyens contre les politiques de dégradation du service public. Je pense en particulier aux alertes émises par le CHSCT de la SNCF sur l'état des voies ferrées de Brétigny, dont on connaît les conséquences tragiques. Si les atteintes au droit fondamental à la santé ont pu être dénoncées, c'est en grande partie grâce aux CHSCT, qui ont un rôle spécifique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et qui disposent de prérogatives importantes, comme les droits d'alerte et d'expertise. La volonté du Gouvernement- neutraliser l'action de ces comités -n'est finalement qu'une réponse apportée au patronat et aux directions administratives de la fonction publique. Ces derniers désirent mettre un frein à l'expression collective des salariés sur leurs conditions de travail, en réduisant le nombre des représentants de ceux-ci, leurs moyens, et en les éloignant des collectifs de travail. C'est ce que l'on observe déjà dans le secteur privé avec la mise en place des comités sociaux et économiques, les CSE, depuis 2017. À cet égard, une note d'étape d'évaluation de l'ordonnance relative au dialogue social, élaborée par France Stratégie, relève que la mise en place des CSE est dominée par un souci de rationalisation économique, et qu'elle n'a pas renouvelé la dynamique du dialogue social. Tel est, précisément, l'unique objectif de la fusion des instances : faire des économies sur la représentation des

des améliorations significatives des conditions de travail. Par leur faculté d'enquête et de visite de sites, ils ont contribué à améliorer les dispositifs de prévention et à faire reculer, dans de nombreuses administrations, les risques de souffrance au travail. Ils sont le lieu idéal pour mettre en oeuvre les dispositifs de lutte contre les violences sexistes pour prévenir, identifier et résorber les situations de harcèlement ; pour prendre en compte, de manière générale, la santé des agents au travail. Les CHSCT permettent à la fois d'améliorer les conditions de travail des agents et d'informer, et donc de protéger l'employeur, dont la responsabilité peut être engagée en cas d'absence de réponse et d'anticipation des risques de harcèlement notamment. Qu'en sera-t-il à l'heure des réorganisations de services, avec les situations de gestion du stress qui en découleront ?

que « le retour [ ...] à une instance unique aurait comme conséquence d'affaiblir et de diluer le travail à mener sur des thématiques très différentes et dont l'importance justifie une approche et des moyens

ne va rien changer, sauf pour la disponibilité et la compétence des délégués du personnel, qui, depuis 2014, se sont spécialisés pour répondre aux problématiques d'hygiène, de sécurité et de santé.

ne va rien changer- et c'est bien dommage -quant à la lutte contre la souffrance au travail, qui est un véritable fléau, à la prévention des burn-out, encore non reconnus, et au signalement des problèmes de santé de très nombreux agents- je pense en particulier à la fonction publique hospitalière,

bien d'une remise en question du dialogue social dans notre fonction publique. J'insiste sur la spécificité des CHSCT,

personnellement les hommes et les femmes qui exercent des missions de service public. Alors que le Gouvernement prépare des restructurations importantes dans la fonction publique, cette proposition de fusion, qui conduit- admettons-le ! -à la disparition de cette structure, est un mauvais signal et un lourd motif d'inquiétude.

dans le cadre de ses fonctions. Sur la question de la représentativité, les comités sociaux d'administration, d'établissement ou territoriaux, seront élus à l'occasion des élections professionnelles de 2022.

mais de l'amélioration de l'offre, du choix des opérateurs, de l'information, du coût, de la qualité, des modalités et de la stratégie du service public. Comment parler de stratégie

vise à garantir que les comités sociaux seront informés des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois. Les comités techniques sont actuellement consultés sur ces questions, conformément à l'article 15

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a introduit un dispositif en vertu duquel un employeur public, pour des fonctions nécessitant une qualification technique spécialisée, peut bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'employeur public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés. Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

est reconnu dans le secteur privé depuis le 1 janvier 2017, en application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. la problématique du droit à la déconnexion n'est pas propre aux salariés du secteur privé ; l'apparition des outils numériques et leur usage dans la vie professionnelle ont aujourd'hui des conséquences importantes sur la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents ainsi que sur le respect des temps de repos et de congé. En pratique, les comités sociaux seront désormais consultés sur les modalités d'exercice de ce droit à la déconnexion et de mise en oeuvre des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. Nous souhaitons donc que cela soit explicitement inscrit dans le texte.

l'affirmation d'un droit à la déconnexion dans les termes que vous proposez ne serait pas aisément compatible avec certaines obligations de service, de continuité et d'astreinte. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour l'obligation de travailler sur les enjeux

vote. Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'État, de ne pas être d'accord avec votre argumentation. On ne peut pas tout mélanger : le statut de la fonction publique impose, certes, aux fonctionnaires des obligations, parmi lesquelles celle d'assurer la continuité du service public, et des outils sont prévus à cet effet.

L'amendement que nous proposons vise, quant à lui, à faire bénéficier les agents du droit à la déconnexion, c'est-à-dire du droit de ne pas être pollués dans leur vie privée par des mails intempestifs qui, dès lors

À défaut du maintien des CHSCT, cet amendement de repli fixe à cinquante agents le seuil à partir duquel il serait obligatoire de mettre en place, au sein des comités sociaux, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Kern. La poursuite des politiques et de l'action des centres de gestion en matière de prévention pour la santé et la sécurité au travail justifie que les projets puissent être poursuivis dans le cadre de la nouvelle formation spécialisée, dont la création permettra aux collectivités et établissements de disposer d'une instance auprès du centre de gestion, qui poursuivra ainsi l'action de l'ancien CHSCT. Les deux amendements

l'idée d'une coconstruction du texte avec les représentants des employeurs territoriaux. Dans la mesure où, par courrier, l'Association des maires de France a ouvertement et formellement pris position pour le seuil de deux cents ETP et que celui-ci a été repris

parlementaires qui se sont exprimés sur le sujet et les organisations syndicales. Cette incompréhension porte sur l'importance croissante des problématiques de santé, d'hygiène et de sécurité dans l'ensemble du monde de travail.

à la complexité croissante des procédures, le tout provoquant de plus en plus de souffrance au travail. Or nous avons la conviction que

elle pourrait être saisie par un certain nombre de comités sociaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. De fait, pour l'avoir vécu dans un passé relativement lointain, je me suis bien rendu compte que les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail

Le projet de loi prévoit que la formation spécialisée ne sera pas consultée lorsque les questions de santé, de sécurité ou d'organisation du travail se posent dans le cadre de « projets de réorganisation de services

sur le procès des responsables de France Télécom qui avaient engagé une très vaste réorganisation de leurs services, avec les conséquences que l'on connaît. Nous avons cru comprendre

important de maintenir l'avis des formations spécialisées en cas de réorganisation de services.

Or cette disposition permettra aux comités sociaux de s'exprimer de manière globale, sans risque que plusieurs formations spécialisées ne se contredisent sur un projet de réorganisation qui les concerne. Cette précision nous semble plutôt favorable aux agents, car elle permet que leurs représentants s'expriment clairement sur un sujet donné. L'avis est donc défavorable.

sincèrement, nous pensons que le niveau de technicité nécessaire aujourd'hui pour aborder les questions de santé, les risques psychosociaux et toutes les problématiques d'hygiène et de sécurité est tel qu'il nécessite des délégués très spécialisés.

parmi les représentants élus au comité social. Les représentants titulaires ont donc toute la légitimité de l'élection, et les organisations syndicales peuvent les choisir parmi les élus ; elles peuvent aussi présenter aux élections des personnes hautement qualifiées,

Instituer deux suppléants par titulaire reviendrait, dans les faits, à permettre aux organisations syndicales de faire plus facilement siéger des représentants qu'elles auraient librement choisis et qui n'auraient pas été élus par les agents. De mon point de

Les compétences requises au sein d'un comité technique et celles requises au sein d'un CHSCT ne sont pas les mêmes. Au fur et à mesure des années, depuis que les CHSCT existent dans la fonction publique, les délégués du personnel se sont spécialisés pour répondre à des problématiques de plus en plus aiguës.

que pour les employeurs, car la prévention des risques de santé, en particulier des risques de harcèlement, protège les uns et les autres. On se démunit en réduisant la capacité des délégués du personnel à intervenir comme ils l'ont fait

de l'existence et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseil exerce les compétences des comités techniques et celles du futur comité social d'administration pour les questions touchant les magistrats, tandis que celles touchant les agents des greffes relèvent d'un comité technique au sein duquel les magistrats ne sont pas représentés. L'amendement vise à maintenir l'existence d'une instance reprenant les compétences de l'actuel comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et regroupant des représentants des magistrats des magistrats et des agents des greffes pour connaître des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Si, aux termes de l'article 33 de la loi de 1984, le rapport présenté au comité technique dresse notamment le bilan des recrutements, des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel, la réécriture de ces dispositions par l'article 3 du présent projet de loi ne reprend pas ces précisions. L'Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire, au motif que ces données seront comprises dans les lignes directrices de gestion. Il s'agit à nos yeux d'un contresens, puisque les lignes directrices de gestion détermineront des orientations générales sur la base du rapport social unique. C'est donc bien ce qui doit rassembler les données relatives aux recrutements, aux avancements, aux actions de formation et aux demandes de travail à temps partiel et de télétravail, ainsi qu'aux demandes de mobilité. Sur la base de ces données, l'autorité territoriale déterminera les lignes directrices de gestion. Nous souhaitons donc remettre les choses à l'endroit

En l'état actuel du droit, les représentants syndicaux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l'exercice de leur droit syndical d'un crédit de temps syndical comprenant deux contingents : un contingent d'autorisations d'absence et un contingent de décharges d'activité de service.

notre amendement est quasi identique à celui du Gouvernement. La commission des lois a remplacé le crédit de temps syndical accordé aux représentants du personnel qui siègent dans les comités sociaux territoriaux par des autorisations spéciales d'absence, sur la base de considérations exclusivement budgétaires. Outre que l'exercice des droits des syndicats ne peut s'envisager sous ce seul prisme, le régime des autorisations spéciales d'absence est plus restrictif

Le crédit de temps syndical correspond à un volume d'équivalents temps plein représentant une charge obligatoire pour les centres de gestion. Nous préférons la solution moins onéreuse consistant à autoriser un représentant du personnel à s'absenter pour exercer sa mission. Avis défavorable sur les deux amendements.

les moyens dont disposent les organisations syndicales au titre de leur représentativité pour exercer leur mandat. Si nous accompagnions la réforme d'une règle purement arithmétique, une règle de trois, la diminution des moyens serait telle que les conditions et les capacités d'exercice des fonctions syndicales non par les délégués, mais par les organisations syndicales elles-mêmes, seraient extrêmement compliquées, voire précaires. Nous avons pris l'engagement d'une concertation, puisque nous traitons ce sujet par voie réglementaire. Vous proposez de limiter le champ d'action du pouvoir réglementaire aux seules autorisations d'absence, ce qui nous paraît trop contraignant à ce stade. Nous souhaitons trouver le bon équilibre entre la mise en oeuvre de la réforme, avec une diminution du nombre d'instances, et les moyens dont peuvent disposer les organisations syndicales pour exercer pleinement leurs droits, leurs fonctions et leurs responsabilités auprès des agents et dans les instances. C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister pour

secrétaire d'État. Votre commission des lois a souhaité élargir le périmètre des compétences du comité social d'établissement des établissements publics de santé à la question de l'autonomie et de l'offre de santé, alors que les dispositions initiales concernaient l'offre de soins.

Nous ne souhaitons donc bien évidemment pas qu'elle soit remise en cause. L'offre de soins n'inclut pas les politiques en faveur de l'autonomie. Or il est nécessaire de le préciser. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre l'amendement du Gouvernement.

: La parole est à M. le secrétaire d'État. Cet amendement vise à clarifier le fait que le comité social d'administration du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas compétent pour l'examen des questions statutaires des corps des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur.

en commission, sur l'initiative de M. Marie. Selon le Gouvernement, la formulation retenue par la commission est plus large que les attributions des établissements auprès desquels sont placés les comités sociaux. Il semble naturel que, parmi ces politiques, le comité social ne se penche que sur ce qui relève de l'établissement dont il dépend. Une formulation un peu plus large n'est donc pas pénalisante et évite de laisser des angles morts dans la définition des compétences. En conséquence, l'avis est défavorable.

de la représentation du personnel de La Poste, dans l'attente d'évolutions à l'issue des prochaines élections professionnelles prévues à la fin de l'année 2022. L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a abrogé les dispositions légales relatives aux comités d'entreprise et aux CHSCT au fur et à mesure de l'organisation des élections professionnelles dans les entreprises et, au plus tard, au 1 janvier 2020,

pour lesquelles des ambiguïtés demeurent après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise. L'amendement prévoit explicitement que les dispositions du code du travail relatives aux CHSCT et qui sont antérieures à cette ordonnance seront maintenues en vigueur pour ce qui concerne La Poste jusqu'au prochain renouvellement des instances et jusqu'à la mise en place d'un comité social d'établissement. L'avis est donc favorable.

il l'est, d'une part, pour les nombreux fonctionnaires ultramarins présents dans l'Hexagone qui attendent souvent des années un retour qui ne vient jamais et qui ne comprennent pas toujours les refus à leurs demandes de mutation il l'est, d'autre part, pour les territoires d'outre-mer, car le retour de leurs forces vives est devenu une nécessité. C'est particulièrement le cas pour la Martinique et la Guadeloupe, seules régions de France à perdre massivement des habitants. La Martinique, par exemple,

des différentes fonctions publiques dans ces collectivités. Ainsi, cet amendement vise à consacrer un chapitre du rapport social unique à la question des mutations et détachements de fonctionnaires vers les collectivités dites d'outre-mer. Il permettra de mesurer l'évolution de ces mutations de façon transparente et d'objectiver les efforts qui doivent être réalisés en la matière. Quel

pour les administrations situées outre-mer qui souhaitent enrichir leur rapport social unique à ce sujet, les éléments et les données demandés. Cette question, qui représente un enjeu important pour les agents ultramarins, sera de nouveau abordée lors de l'examen des articles 11

secrétaire d'État. Les députés, sur l'initiative de leur rapporteur, ont voulu simplifier les conditions du dialogue social, notamment en créant un rapport social unique. Votre commission, qui s'est saisie de cette proposition, a apporté un certain nombre de modifications ; je pense notamment à la question de la périodicité et de la publicité du rapport.

il tend à retirer du rapport social unique le bilan de la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, qui, à notre sens, doit demeurer autonome : c'est là l'un des principaux changements que nous apportons au dialogue social. il prévoit d'ajouter les effectifs au contenu du rapport social unique, d'associer la diversité et la lutte contre les discriminations, deux notions étroitement liées, et de fondre dans la mobilité les éléments de mise à disposition en vue d'avoir une lecture plus cohérente. Quatrièmement, il vise à enlever les éléments qualitatifs du rapport qui n'ont pas à se retrouver dans la base de données, ainsi que les périodes sur lesquelles portent les données accessibles. Cinquièmement, la présentation de ce rapport devant les assemblées délibérantes pour le versant territorial de la fonction publique dans la mesure où celui-ci fera l'objet d'un examen au sein du comité social. Chaque élu sera de le présenter ou non- nous en débattrons -à son instance délibérante. Sixièmement, nous souhaitons rétablir les articles relatifs aux rapports sur les mises à disposition et les mutilés de guerre et assimilés, des informations qui nous semblent importantes, même si elles ne concernent évidemment pas tous les établissements publics.

contre le harcèlement moral au sein de la fonction publique parmi les éléments constitutifs du rapport social unique tel qu'il est défini par le présent article. Le harcèlement moral est un délit qui entraîne pour celui qui en est l'objet la dégradation des conditions de travail, la dépression et un risque de maladie physique ou mentale en relation avec l'épuisement professionnel, le burn-out. Toutes les administrations avaient l'obligation, en liaison avec les représentants du personnel et, s'il existe, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral. Pour ce faire, ce dernier disposait d'un droit d'alerte, qui lui permettait de prévenir l'administration de tout cas de harcèlement moral. Avec le présent projet de loi, en prévoyant la fusion des comités techniques et des CHSCT au sein d'une structure unique qui prend le nom de « comité social », il apparaît indispensable d'introduire clairement, au moins dans le cadre du rapport social unique, la prévention et la lutte contre le harcèlement moral

Concernant l'amendement n° 326, le Gouvernement a assoupli quelque peu sa position, notamment sur la périodicité du rapport social unique. Il accepte le caractère biennal, mais renvoie à un décret la possibilité de prévoir une périodicité plus courte. Je vous propose, en attendant la réunion de la commission mixte paritaire, de nous en tenir à la rédaction adoptée

et données du rapport social unique. Ce dernier intègre dans l'état de situation comparée des données sexuées relatives aux actes de harcèlement moral. Peut-être faut-il le faire apparaître plus clairement. Aussi, la commission s'en remet à la sagesse

entre les femmes et les hommes, tout comme les données relatives aux violences sexuelles et sexistes qui incluent, en application de l'accord du 30 novembre 2018 dans la fonction publique, le harcèlement sexuel et moral. En conséquence, votre demande est satisfaite.

vise à préciser le contenu du rapport social unique en indiquant qu'il devra intégrer les éléments et données relatifs aux avancements, qui en ont été écartés. Or cela nous paraît fondamental pour l'information des partenaires sociaux. Quel

d'arrêt maladie. Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l'information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, 56 % des collectivités territoriales seulement participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance. C'est pourquoi nous proposons de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l'acquisition d'une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

Cette situation, ajoutée au rétablissement, en 2018, du jour de carence, se traduit par une augmentation de la durée et de la fréquence des arrêts de travail et un fort absentéisme. Or les agents publics territoriaux sont soumis à des conditions de travail difficiles et sont exposés à des risques professionnels importants.

Enfin, 12,5 % d'entre eux travaillent la nuit. La situation risque donc de se dégrader, ce qui induit de lourdes conséquences pour les collectivités, les agents, ainsi que les usagers. Dans ce cadre, la protection sociale complémentaire des agents territoriaux constitue un enjeu double en termes d'intérêt général : un enjeu en matière de santé publique pour 1,9 million d'agents territoriaux matière de pouvoir d'achat pour ces agents, dont 75 % appartiennent à la catégorie C et peuvent tomber sous le seuil de pauvreté en cas d'arrêt de longue durée s'ils ne sont pas couverts au titre Ces derniers sont moins bien protégés que 85 % des salariés du privé, qui bénéficient d'une couverture prévoyance obligatoire et financée par leur employeur. À la différence du secteur privé où la participation des employeurs à l'acquisition d'une complémentaire santé est obligatoire, celle-ci reste facultative dans la fonction publique, notamment de santé des agents territoriaux est d'autant plus préoccupante que, dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d'arrêt maladie, ce qui complique alors un durable retour à l'emploi dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, seulement 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance. Dans l'intérêt des agents publics et des usagers du service public local, cet amendement vise à assurer aux agents publics un haut niveau de prévention, de santé et de protection sociale, en introduisant dans le rapport social unique, qui est destiné à être le document de pilotage du bilan ressources humaines dans les collectivités et qui sera présenté en assemblée délibérante, le sujet de l'accès et du financement de la complémentaire santé et de la prévoyance. La parole est à Mme Corinne

Les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient ainsi augmenté de 26 % entre 2007 et 2015. L'aggravation de l'état de santé des agents territoriaux est d'autant plus préoccupante que cette population n'a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d'arrêt maladie, ce qui complique alors un retour à l'emploi durable dans de bonnes conditions. Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l'information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, comme cela a été souligné à deux reprises, seulement 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance. C'est la raison pour laquelle notre amendement tend à compléter le rapport social unique que crée crée cet article. Certes, ce rapport social unique introduit plus de cohérence entre les politiques de ressources humaines des collectivités territoriales, mais il présente des limites. Il ne s'agit là que d'un bilan social, qui permettra d'éclairer les élus locaux sur la situation de leurs agents, en fonction de leur volonté, et n'engage donc pas de décision concrète. Ce rapport ne sera pas soumis à délibération, mais il sera uniquement rendu public. Les enjeux liés à la protection sociale complémentaire des agents publics ne sont pas explicitement intégrés à ce stade dans ce bilan.

L'article 3 A du projet de loi prévoit que les administrations établissent chaque année un rapport social unique, qui servirait de base pour l'élaboration des lignes directrices de gestion. Celui-ci comprendrait des informations relatives au recrutement, à la formation ou encore aux parcours professionnels des agents publics. L'amendement qui vous est présenté vise à inclure au sein dudit rapport des informations relatives aux aides à l'acquisition d'une protection sociale complémentaire santé et prévoyance, notamment Rassurez-vous, l'objet de cet amendement est non pas d'aboutir à un inventaire à la Prévert des données comprises dans le rapport social unique, mais bien de répondre à une problématique empiriquement constatée dans les administrations, et plus particulièrement au sein des collectivités territoriales. En effet, si l'amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents contribue pleinement à une qualité accrue du service public, force est de constater le sentiment de dégradation du bien-être au travail que ressentent les deux tiers des agents consultés, ce qui se traduit par des conséquences néfastes sur la santé et une du nombre des arrêts de travail dans les collectivités territoriales. Une telle situation est d'autant plus préoccupante que, au sein de la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, notamment chez les plus jeunes, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d'arrêt maladie, ce qui complique alors un retour à l'emploi dans de bonnes conditions. Si la participation financière des collectivités garantit une meilleure information des agents et les incite à se protéger, force est encore de constater qu'elles sont trop peu nombreuses à le faire : seulement 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé, contre 69 % en prévoyance. La mise en place d'un dispositif complémentaire santé ou prévoyance demeure en réalité facultative pour l'employeur public territorial, bien qu'elle soit obligatoire dans le privé. De telles différences ne peuvent être acceptées au regard des inégalités qu'elles créent, Face à une telle situation, l'amendement que je vous présente prévoit de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l'acquisition d'une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

au moyen de la plateforme mise en service à cet effet. Cet amendement a pour objet de tenir compte de l'existant, de l'optimiser et de le mutualiser, d'améliorer et de simplifier l'information et de prendre en compte les investissements financiers et humains très importants qui sont réalisés par les centres de gestion pour mettre à la disposition de l'ensemble des collectivités territoriales une base de données

de la commission ? Ces trois amendements visent à préciser que les centres de gestion rendent accessible un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale. Ceux-ci nous semblent apporter une amélioration tout à fait bienvenue au dispositif en permettant une mutualisation entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Un portail numérique est déjà mis à disposition des collectivités et établissements affiliés par les centres de gestion pour l'élaboration des bilans sociaux. Il est de bonne gestion de pouvoir continuer à utiliser ce portail, au besoin en le faisant évoluer, étant précisé que la direction générale

Mme Christine Prunaud. Alors que l'on constate une dégradation du bien-être au travail des agents territoriaux, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé,

Nous proposons de consacrer un temps de débat des assemblées délibérantes des collectivités territoriales à l'état des lieux et à la stratégie de la collectivité en matière de prévention et d'aide à l'acquisition d'une protection sociale complémentaire, enjeu important de santé publique pour l'ensemble des agents territoriaux. Nous proposons également que ce débat porte tout à la fois sur la protection de la santé physique et mentale, l'hygiène et la sécurité des agents sur leur lieu de travail, l'organisation du travail, l'amélioration des conditions de travail, ainsi que la prévention, l'information et la formation aux risques professionnels. Tout cela est à développer. Il est à nos yeux essentiel que les élus locaux soient tenus informés- afin qu'ils soient davantage impliqués -des conditions de travail des agents de la collectivité, qui assurent au quotidien la bonne marche des services publics de proximité.

sur leur santé. Les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient ainsi augmenté de 26 % entre 2007 et 2015. Les causes de cette dégradation sont diverses : tout d'abord, un contexte marqué par les réorganisations successives du monde territorial avec des transferts de personnels, la mise en place des intercommunalités, les rapprochements entre collectivités et la création de nouveaux syndicats ; ensuite, l'exposition aux risques professionnels physiques- avec 50 % d'agents exerçant des métiers techniques -et aux risques psychosociaux ; enfin, l'accroissement de la moyenne d'âge des agents.

En effet, dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas d'une couverture en prévoyance, si bien qu'il perd la moitié de son traitement après trois mois d'arrêt maladie. Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l'information des agents et les incite à se protéger. C'est pourquoi cet amendement tend à consacrer, tous les trois ans, un temps de débat en assemblée délibérante à la prévention, la santé au travail et aux aides à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. Cette disposition complète le rapport social unique, qui a été introduit à l'article 3 A et dont nous venons de discuter. Si ce rapport social va dans le bon sens en rendant plus cohérente la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales, il n'englobe pas explicitement les politiques de prévention et les aides à la protection sociale complémentaire.

obligatoire sur la protection sociale complémentaire, la protection de la santé physique et mentale, l'hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions de travail, etc.

que la loi du 19 février 2007 rend déjà obligatoire un plan de formation. Seulement, nous constatons tous dans toutes nos collectivités que cette mesure n'est, hélas, pas suffisamment incitative. Nous proposons donc, comme d'ailleurs nous y invite solennellement le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences. Il prévoit également la présentation du bilan de la mise en oeuvre de ce plan lors du débat d'orientation budgétaire de l'assemblée délibérante des collectivités. Dans le cadre du rapport social unique introduit par l'article 3 A, les collectivités locales devront présenter, tous les deux ans, des données relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements et à la formation. Les données du rapport social unique seront en outre le fondement des lignes directrices de gestion, qui détermineront la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Enfin,

à rendre obligatoire la remise d'un nouveau rapport par l'autorité territoriale au comité social territorial. Il s'agirait d'une charge de travail supplémentaire pour les collectivités. Par ailleurs, le champ de ce rapport serait proche, voire très proche, du rapport social unique, lequel contient, sur l'initiative de la commission, une thématique sur la santé et la sécurité au travail. L'absentéisme pourra tout à fait être

Première raison : nous tenons à la démocratie sociale, dans le secteur privé comme dans la fonction publique, et fusionner les différents organes de représentation éloignerait les salariés de leurs représentants et favoriserait la professionnalisation de ceux-ci au détriment d'un dialogue quotidien nécessaire.

la gestion des intérêts communs. Ainsi, le directeur peut réunir conjointement le comité technique et le comité d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel. Le mécanisme proposé ici, qui fusionne les différents comités, complexifierait, je le répète, le fonctionnement des instances de représentation,

Aussi, pour les mêmes raisons qui l'ont poussée à ne pas vouloir supprimer l'article 3, elle ne souhaite pas supprimer l'article 3 , qui étend la solution retenue au cas spécifique des instances de l'Agence nationale de contrôle du logement social. La commission a donc émis un avis défavorable

Par exemple, sur le portail de la fonction publique, il y a une page intitulée « Grilles de carrières de catégorie A+ et divers emplois types de l'administration ». À l'intérieur de cette « catégorie A supérieure on rencontre notamment les administrateurs civils, les architectes et urbanistes de l'État, les professeurs agrégés, les ingénieurs des ponts, des eaux et forêts, mais on peut se demander pourquoi on ne trouve pas mention, par exemple, des ingénieurs des mines. Sur un autre site internet, celui du CNFPT, on trouve une page dédiée à la « préparation aux concours A+

de l'ensemble de la catégorie A, cette catégorie ne sera plus représentée à l'intérieur des CAP, ce qui conduira à un jugement de ces agents non plus par leurs pairs, mais uniquement par leurs collègues. Cela posera un certain nombre de problèmes, notamment au regard de la spécificité des carrières des agents de catégorie A+, et des emplois qu'ils occupent

permettrait de répondre aux lacunes de la gestion des ressources humaines au sein de l'État, Mme Lavarde vient de l'évoquer avec éloquence. Frédéric Thiriez l'a souligné durant son audition, l'État ne gère pas suffisamment ses talents, et la commission d'enquête proposait de créer une véritable DRH de l'État, avec une attention particulière portée aux hauts a rappelé, à l'article 22 du projet de loi, cette exigence de meilleure gestion des carrières. Certes, le chemin est encore long- la mission Thiriez n'a pas encore conclu ses travaux, et identifier le périmètre de la catégorie A+ ne sera pas chose facile -, mais, pour faire avancer les choses, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.

mission, mais il nous semble indispensable d'améliorer fondamentalement la gestion des ressources humaines de la haute fonction publique, et la création de cette catégorie

Assassi, sur l'article. Cet article constitue un grand recul en matière de participation des fonctionnaires aux décisions les concernant. Premièrement, en redéfinissant le périmètre des commissions, qui ne seront plus instituées par corps, mais par catégorie, dans le cadre de la fonction publique d'État, et en supprimant les CAP par sous-groupe hiérarchique au sein d'une même catégorie dans la fonction publique territoriale, le projet de loi déconstruit les collectifs de travail et réduit drastiquement le nombre de commissions, et donc le nombre de représentants du personnel. Deuxièmement, cet article porte atteinte aux prérogatives des commissions administratives paritaires en leur ôtant la possibilité d'intervenir sur les décisions relatives aux mobilités et aux mutations des agents. Le travail effectué en commission

pertinemment que la volonté du Gouvernement de retirer des missions des CAP l'analyse des décisions relatives aux mobilités et aux mutations s'inscrit dans une logique de privatisation de la fonction publique et d'accompagnement des restructurations. Ainsi, c'est l'arbitraire des managers qui est favorisé au détriment des intérêts des personnels. Une fois de plus, vous ne tirez pas les leçons du bilan catastrophique des privatisations et restructurations intervenues notamment chez Pôle emploi,

Mes chers collègues, si nous voulons éviter la reproduction de ces drames, il faut que nous renforcions les prérogatives des instances de représentation au lieu de les détruire comme cela nous est proposé.

désormais traitées la définition, par les employeurs, des lignes directrices de gestion créées par l'article 17 du projet de loi, après consultation des comités sociaux. Toutes les organisations syndicales se sont opposées à cet article et, dans son avis, le Conseil d'État souligne qu'il conviendra de veiller à ce que l'application de cette réforme ne se traduise pas par un appauvrissement du dialogue social. Le constat que l'on peut faire, monsieur le secrétaire est qu'une CAP apaisée est en général à la fois le gage et le signe d'un dialogue social de qualité, qui contribue à l'engagement des agents dans le travail ainsi qu'à leur adhésion à des projets de service et, lorsqu'elles sont nécessaires, à des restructurations., lorsque les choses se passent mal, on peut y voir le symptôme d'un problème plus large. En réalité, les CAP ne sont en rien un problème. Elles sont éventuellement le révélateur de la façon dont les managers- j'emploie ce terme, puisqu'il est consacré -considèrent le dialogue social. D'ailleurs, la volonté qui est la vôtre d'affaiblir les CAP dit également quelque chose de ce que les managers en place au Gouvernement et dans cette majorité pensent du dialogue social et du paritarisme. La simplification serait le parangon de l'efficacité c'est ce même argument qui conduisait le Gouvernement à vouloir réduire les pouvoirs du Parlement. Or ni la démocratie parlementaire ni la démocratie sociale ne sont des choses incommodes dont il faudrait s'accommoder. C'est vrai, c'est long ; mais c'est absolument nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous appelons à la suppression de cet article.

D'autre part, l'évolution de carrière est permise par les pairs, les commissions administratives. Ces règles sont consubstantielles à l'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis de leur hiérarchie, et sont fondées sur le mérite.

Posons par exemple cette question : les fonctionnaires sont-ils au service de la Nation, comme le veut la tradition française, ou vont-ils devenir des dirigeants au moment, comme le veut la tradition anglo-saxonne ? Il y a un choix à faire. Ces attaques, je les connais bien, comme beaucoup d'entre nous. Entre ce projet de loi et celui de votre collègue Jean-Michel Blanquer, c'est la deuxième fois que la question du recrutement et du suivi des carrières des enseignants-chercheurs est posée, par exemple. Le renforcement des pouvoirs des présidents d'université entre pleinement dans la dynamique des réformes Pécresse et Fioraso, qui ont petit à petit affaibli la démocratie universitaire.

d'un examen fondé sur les seuls critères scientifiques. Faire entrer le président de l'université dans le processus, c'est créer un lien hiérarchique entre enseignant-chercheur et président d'université, avec tous les risques que cela peut comporter pour l'indépendance de la recherche et de l'enseignement- d'ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont reconnu qu'un très grand nombre de présidents d'université s'étaient affranchis.

du périmètre d'intervention des CAP, que vous proposez, monsieur le secrétaire d'État, pose de nombreuses questions. Sur des sujets aussi importants dans la carrière d'un fonctionnaire que la mobilité, la mutation, l'avancement, les CAP ne seront plus consultées ; d'une certaine manière, elles deviendront presque exclusivement disciplinaires. Prenons des exemples concrets,

le paritarisme et le travail des syndicats au niveau des corps permettent de réguler ces difficultés dans l'appréciation des barèmes applicables aux demandes de mutation.

la bonne marche des CAP la relation directe entre un chef de service et un agent n'est pas de bonne politique. Nous croyons que le paritarisme est une garantie de transparence et d'équité de traitement,

ce qui est important, les décisions relatives aux mobilités des fonctionnaires- c'est-à-dire les mutations, les détachements, etc. -ne seront plus évoquées dans ces instances de dialogue social. Pourtant, ces instances demeurent absolument essentielles à la vitalité de la démocratie sociale de la fonction publique. Instances paritaires élues au suffrage direct, les CAP constituent des outils prépondérants de dialogue. Dans l'esprit du gouvernement et des parlementaires qui ont instauré ces instances, il s'agissait d'assurer dans le même temps la participation des agents et de l'autorité hiérarchique, afin de protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques. Ces instances permettent ainsi la transparence et donc l'acceptabilité des avis rendus- ce que les lignes directrices du présent projet de loi ne peuvent à elles seules garantir elles protègent contre l'arbitraire. Nous craignons ainsi qu'une telle dévitalisation ne porte le risque d'une conflictualité accrue pour des agents qui ne connaîtront plus les motivations de décisions aux implications pourtant personnellement très engageantes. En procédant de la sorte, le Gouvernement cherche à dupliquer les méthodes du secteur privé dans le secteur public, bien que cette vision aille à l'encontre de la conception républicaine de notre fonction publique et des particularités de sa construction républicaine.

La commission des lois est revenue sur la rédaction initiale de l'article, qui excluait des compétences de la CAP l'ensemble des décisions favorables aux agents. Nous sommes favorables au souhait du Gouvernement d'alléger le fonctionnement des instances, mais avons souhaité réintroduire l'avis des CAP là où il nous semble fondamental, en matière d'avancement et de promotion, notamment. que l'article 4, tel que l'a amendé la commission des lois, est un compromis raisonnable entre simplification, d'une part, et garanties accordées aux fonctionnaires, d'autre part.

va permettre aux employeurs et aux organisations syndicales de délibérer sur le cadre de gestion des ressources humaines, notamment sur les règles générales d'accès à la mobilité et à la promotion.

Nous considérons que ces règles d'accès à la mobilité, à la promotion, seront rendues publiques et que, ce faisant, le barème y afférent sera tout aussi public, ce qui permettra de faire la transparence sur les critères de choix. Les CAP resteront compétentes pour d'autres sujets que les sujets disciplinaires : elles demeureront évidemment compétentes pour rendre un avis préalable en matière disciplinaire, en matière d'insuffisance professionnelle, en cas de refus de titularisation, de licenciement en cas de refus de trois postes successifs pour un fonctionnaire placé en disponibilité demandant sa réintégration, de refus de congé de formation syndicale, de refus de formation, de congé de formation professionnelle, ou encore en cas de déchéance ou de restriction du droit à pension. Par ailleurs, elles interviendront en tant qu'instance de recours à la demande de l'agent sur les décisions individuelles défavorables autres que celles qui sont liées aux mobilités ou, dans la version du texte du Gouvernement, aux promotions et avancements, puisque ces décisions-là feront l'objet d'un recours spécifique.

L'exercice de ces prérogatives exorbitantes liées au statut, qui crée d'abord des obligations pour les fonctionnaires, se fait sous le regard non décisionnel des partenaires sociaux. Dans le moment que nous vivons, je crois, monsieur le secrétaire d'État, non pas à une forme plébiscitaire d'exercice du pouvoir à tous les niveaux, y compris au niveau local, mais, inversement, à une démocratie sophistiquée dans ses procédures, qui reconnaît le pouvoir des contre-pouvoirs et des organisations syndicales. Je ne vois pas en quoi la réduction du périmètre des CAP, telle que vous la concevez, améliorera le dialogue social. Bien au contraire, il s'en trouvera

tout en conservant le bénéfice d'une aide en cas de recours administratif. Mais, hélas, ce n'est pas suffisant : nous savons ce que représentaient historiquement les CAP comme contrepartie pour les fonctionnaires, qui ont des obligations statutaires, comme vient de le rappeler mon collègue Didier Marie. Soustraire au regard des des partenaires sociaux des éléments relevant de la gestion des carrières et de l'application des règles du statut trouve évidemment un écho dans le recours considérablement accru aux contractuels, qui, précisément, ne se trouvent pas dans cette situation statutaire. Nous aurions pu concevoir que, sur la base d'un diagnostic partagé, on modernise les CAP, mais tel n'est pas le cas, puisque celles-ci sont affaiblies de manière inédite. Et puisque ceux qui proposent cette réforme proclament leur amour du dialogue social, je leur rappellerai que les neuf organisations syndicales sont opposées à cette disposition. Dernière remarque : la liste des attributions des CAP sera désormais établie par décret en en Conseil d'État, alors que cela se faisait auparavant uniquement par la loi. Il est donc demandé aux parlementaires de légiférer à l'aveugle, alors que le Gouvernement s'était engagé à présenter les projets de décret en même temps que le projet de loi.

au sein de chacune des catégories et, d'autre part, à la diversité d'emplois que peut recouvrir chaque catégorie. Cette proposition va créer de la confusion, alors que, aujourd'hui, les choses fonctionnent plutôt bien.

Le fait que puissent être créées « une ou plusieurs » CAP par catégorie conduira à redécouper les catégories à l'intérieur de chaque structure de l'administration de l'État. Il est fort probable que ce redécoupage se rapproche, de fait, du découpage par corps existant.

l'avis du Gouvernement ? Il est défavorable puisque, comme l'a laissé entendre Mme la rapporteur à l'instant, l'article 4 laisse la possibilité d'instituer une ou plusieurs CAP par catégorie. Il sera donc possible de distinguer plusieurs univers au sein d'un même ministère ou au sein d'un même service, par exemple, au sein du ministère de l'éducation nationale, entre les corps enseignants et non enseignants, même si je sais que cette présentation est par trop réductrice. L'objectif est de pouvoir prendre en considération les différentes filières au sein des administrations, ainsi que les sujétions particulières induites par certaines professions.

par catégories, sans compter la déclinaison par corps. Je veux bien retirer cet amendement au bénéfice du doute, considérant que et le Gouvernement et le rapporteur y sont opposés. Mais je crains que cet article ne contribue pas à la simplification des procédures.

en cas d'examen de nature disciplinaire. Ces dispositions nous semblent être des dispositions de nature réglementaire. Par ailleurs, je viens d'indiquer que nous considérons comme possible qu'un certain nombre d'agents d'agents participent, comme nous l'ont demandé certaines organisations syndicales et les employeurs territoriaux notamment, à l'évaluation de la situation d'agents pouvant appartenir à un autre groupe hiérarchique que le leur.

La combinaison de ces deux dispositions fait que, dans certains cas, tous les représentants du personnel d'une CAP commune ne pourront pas s'exprimer. Nous avons donc introduit, en commission, un mécanisme permettant de garantir la parité de la CAP en diminuant, en proportion, le nombre de représentants de l'employeur public.

Nous considérons que les agents peuvent participer à l'évaluation d'agents de catégorie inférieure. Cela conduirait à maintenir la composition de la CAP sans avoir à la réduire en fonction de la catégorie à laquelle appartient celui ou celle qui fait l'objet d'une sanction potentielle.

On le sait, derrière cet argument, on retrouve l'idée que, en gagnant du temps, on fait des économies bien utiles dans un contexte global d'assèchement des finances publiques. Nous craignons pourtant tout l'inverse. En privant des instances paritaires de prérogatives, vous risquez de gripper la machine, de renforcer la conflictualité, de susciter les incompréhensions et donc, on le répète, la suspicion d'arbitraire. Tout cela risque de créer au final un sentiment de crispation sociale qui n'est favorable ni à la fluidité ni à la bonne marche du service public. Certes, la majorité de ces décisions sont positives, comme vous le rappelez, mais le risque porte sur les 10 % à 20 % de cas défavorables : les agents concernés auront eu le sentiment, au travers de cette réforme, non seulement de ne plus être représentés par une organisation syndicale, mais également que, potentiellement, la décision défavorable est injuste. Cet amendement, à l'inverse de la vision portée par le Gouvernement, tend donc à imposer non pas un renvoi article par article, mais bien un principe général de consultation des commissions administratives paritaires sur l'ensemble des décisions individuelles, et ce, pour l'ensemble des trois fonctions publiques. Il s'agit ainsi

Mme la rapporteur l'a dit il y a un instant : la commission des lois du Sénat a souhaité restaurer la compétence des CAP en matière de promotion et d'avancement ; le Gouvernement considère que le retrait des compétences des CAP en matière de mobilité-mutation et de promotion-avancement s'inscrit dans cette entreprise de simplification que nous recherchons. Nous considérons, comme je le disais il y a un instant en réponse aux intervenants sur les amendements de suppression de l'article, que la définition des lignes directrices de gestion et la définition des règles de mobilité et des règles de promotion par le comité social d'établissement d'administration territoriale, avec la publicité des barèmes- fonction et conséquence de ces règles générales d'accès à la mobilité ou à la promotion -, répondent à la demande de simplification, de transparence et de plus grande confiance témoignée envers les encadrants et les employeurs locaux, qu'ils soient territoriaux ou d'État. Beaucoup souhaitent cette autonomie, nous souhaitons leur faire confiance et leur donner cette autonomie, et nous souhaitons qu'elle puisse s'exercer en matière de mobilité, mais aussi en matière de promotion et d'avancement et donc de gestion des équipes, de management des services et des ressources humaines. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite du Sénat le rétablissement des dispositions supprimant l'examen des dossiers individuels de promotion ou d'avancement

est à M. Arnaud de Belenet. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la suppression de la compétence des CAP pour les mutations à l'intérieur d'une même collectivité ou d'un même établissement comportant un changement de résidence administrative.

Ces sujets sont suffisamment importants pour les agents pour qu'ils soient soumis à l'avis des CAP, gage d'une procédure transparente garantissant effectivement les droits des fonctionnaires, notamment celui d'être représentés.

compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, les mêmes restrictions que celles qui sont prévues à l'article 4 pour les commissions administratives paritaires.

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 4 , qui étend les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues à l'article L. 953-6 du code de l'éducation à l'ensemble des corps des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, en incluant désormais les corps sociaux, de santé et de bibliothèques.

secrétaire d'État. Il s'agit d'appliquer les dispositions relatives à la réforme des CAP à l'établissement public industriel et commercial Universcience, dans la même logique de déploiement que d'autres amendements précédemment présentés.

secrétaire d'État. En l'état actuel du droit, les collectivités territoriales et les établissements publics issus d'un regroupement, d'une fusion ou nouvellement créés sont déjà tenus de définir, après consultation du comité social territorial, si l'on prend le nouveau terme, les régimes indemnitaires applicables à leurs agents dans un délai raisonnable. Ce délai est parfois fixé par le législateur, comme dans le cadre du regroupement des régions, en vertu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. à titre individuel, les agents bénéficient d'un certain nombre de garanties, que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause. Ainsi, nous ne voulons pas remettre en cause l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui ne permet pas de reprendre un avantage collectif existant avant 1984, mais qui permet aux agents transférés à titre individuel de continuer à en bénéficier. À l'inverse, les régimes de travail ne sont pas considérés comme un avantage acquis transférable. Il appartient donc à la nouvelle entité de fixer une organisation du temps de travail dans le respect des règles de droit commun. Cet amendement tend donc à supprimer des dispositions adoptées par votre commission des lois, dont celle qui soumet les collectivités ou les établissements créés

des agents dans un délai de deux ans suivant la création, le regroupement ou la fusion de services de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux. Nous avons tenté de mettre en place ce dispositif. Mais des contraintes induites et des difficultés techniques

Au fil des consultations, puis de la réunion des instances de représentation des agents publics et des employeurs territoriaux est apparue une demande portée notamment par une organisation syndicale, la CFDT, sur l'opportunité de de permettre aux employeurs territoriaux ou aux chefs de services déconcentrés de négocier des accords locaux majoritaires avec leurs organisations syndicales. Les champs d'une telle discussion et de la possibilité de conclure des accords locaux doivent être définis. Il est bien évident certain nombre de champs fondamentaux, comme le profil de rémunération des agents publics à l'échelle d'une carrière ou le temps de travail que nous voulons fixer par la loi de manière aussi uniforme que possible à l'échelon national, ne peuvent pas relever d'un accord majoritaire local.

d'accord national, les acteurs locaux du dialogue social puissent conclure un tel accord avec des règles de validation conformes à ce que nous appelons communément les « règles de Bercy », qui avaient fixé le cadre des accords majoritaires dans la fonction publique.

locaux. Ensuite, nous avons besoin d'un peu de temps pour définir les champs dans lesquels ces accords majoritaires pourraient être d'abord discutés, puis appliqués. La concertation prévue pour rédiger l'ordonnance nous permettra d'en disposer.

de l'Assemblée nationale et du Sénat. Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le rétablissement de l'article 5, habilitant à légiférer sur le dialogue social de proximité et la possibilité d'accords majoritaires locaux.

dans la fonction publique, nous refusons que le Gouvernement légifère par ordonnances sur un sujet aussi important, d'autant plus qu'aucune disposition législative n'a jamais conféré de valeur normative aux accords négociés avec les représentants des agents publics. Comment ne pas voir que cet article s'inscrit dans le droit fil des ordonnances Travail, dont les principes sont désormais appliqués aux emplois publics ? Par conséquent, au-delà des ordonnances, il me semble extrêmement important d'obtenir des clarifications sur l'articulation entre les différents niveaux de négociation. À nos yeux, il faut impérativement maintenir le principe de faveur, selon lequel aucun accord local ne peut être moins favorable aux agents qu'un accord national.

Une des causes principales de ce retard réside dans le fait que l'initiative de la négociation est aujourd'hui exclusivement réservée à l'administration. Dans le secteur privé, les articles du code du travail définissent les thèmes qui sont soumis à une négociation annuelle obligatoire. Au-delà de ces sujets, ce sont les conventions collectives qui prévoient les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. Dans la fonction publique, c'est seulement dans le cas d'un préavis que les parties intéressées « sont tenues de négocier sur les motifs du recours à la grève

Cela nous semble une ouverture utile. Le dialogue social est toujours préférable au conflit, à moins de vouloir organiser le conflit pour des raisons de stratégie politique. Mais je n'ose penser que ce soit cela qui vous anime

La grève, la grève, la grève, ou rien du tout ! » Je ne suis pas sûr, quelle que soit la majorité, que

Mme Christine Prunaud. Cet amendement est très simple. Alors qu'il existe dans le privé un régime de sanctions spécifiques réprimant l'entrave à la liberté et au droit syndical, un tel dispositif n'existe pas pour la fonction publique. Pourtant, pour les salariés du privé comme pour les fonctionnaires, la liberté syndicale est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Il s'agit d'une liberté universelle proclamée par les traités internationaux, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. À l'inverse, dans la fonction publique, les administrateurs d'un syndicat professionnel peuvent faire l'objet de poursuites pénales au titre de l'article L. 2136-1 du code du travail.

en renvoyant, pour ce type de délit, aux sanctions prévues par l'article 432-1 du code pénal, soit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Nous savons que la justice administrative est compétente pour sanctionner de tels agissements, notamment au titre de l'article 8 de la loi du 13 Pour autant, nous souhaitons qu'il soit clairement indiqué que des sanctions pénales et non pas simplement administratives peuvent s'appliquer à de tels agissements.

Cet article garantit le droit syndical et prévoit que les organisations syndicales peuvent ester en justice. Le renvoi à ces dispositions larges et l'utilisation du terme « faire échec » ne permettent pas de définir avec suffisamment de précision les actes matériels qui sont incriminés. Le principe constitutionnel de précision de la loi pénale n'est donc pas respecté. Pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement. Quel est partage l'avis de la commission. Au demeurant, les dispositions applicables à l'heure actuelle permettent à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre toutes mesures permettant d'éviter que des activités ayant un caractère illicite ne portent atteinte au bon fonctionnement des organismes de consultation

la protection des délégués du personnel et des autres instances représentatives au sein de la fonction publique. L'objectif est de donner les mêmes droits aux délégués du personnel dans le secteur privé et dans la fonction publique.

Aussi, pour redonner tout son sens au principe de participation dans la fonction publique et restaurer la confiance des agents dans ce principe, nous proposons, comme à l'amendement précédent, de renvoyer les entraves aux instances de représentation du personnel au régime de sanctions prévu à l'article 432-1

il tend à opérer un tel changement de degré dans la place des contractuels qu'il induit nécessairement un changement de nature de l'ensemble de la fonction publique. de la fonction publique. Le recours aux contractuels, qui sera au coeur des amendements que nous allons examiner, sera central dans cette évolution. Le projet de loi tend à multiplier les possibilités de recourir aux agents contractuels dans toutes les catégories d'emploi des trois fonctions publiques, en particulier pour la quasi-intégralité des postes de direction.

La plupart des dispositions du projet de loi permettent de contourner le statut en multipliant les possibilités dérogatoires de recruter les agents publics par la voie du contrat, en expérimentant la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires ou en contraignant les fonctionnaires à être détachés d'office auprès d'organismes privés, sous la forme d'un CDI en cas d'externalisation de leur service ou de leur mission.

Les quantités de possibilités qui sont offertes de recourir aux contractuels sont réellement de nature à miner le statut

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Il n'est pas question de « vieux monde », c'est un principe fondateur

Depuis lors, le concours est devenu la voie d'accès à ces emplois. En permettant un recours accru aux contractuels dans la fonction publique, le projet de loi tourne le dos à la conception française de la fonction publique de carrière au profit de la fonction publique d'emploi, organisant une administration aux ordres et donc inféodée au pouvoir politique. Il organise parallèlement la précarisation des agents publics, car les contractuels n'ont bien sûr pas les mêmes droits que les fonctionnaires. Une telle conception porte atteinte, notamment pour la fonction publique territoriale, à la continuité de l'action publique. D'ailleurs, les maires ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont vu dans ces dispositifs non pas une opportunité d'élargir le vivier, comme le Gouvernement le préconise, comme le Gouvernement le préconise, mais un risque de déstabilisation de l'ensemble de l'administration et des services publics locaux, créant par là même de grandes inégalités territoriales. En effet, la contractualisation de la fonction publique prévue par le Gouvernement produira un certain nombre d'effets néfastes comme le retour du clientélisme et de la corruption. La contractualisation va aggraver la précarité statutaire de ces nouveaux personnels, mais aussi les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Certes, il est prévu que

Le Quai d'Orsay a vu ses effectifs fondre de 53 % ces trente dernières années, dont un tiers depuis 2008. Aujourd'hui, le Gouvernement annonce encore la suppression de 10 % des personnels actuels dans le cadre du plan Action publique 2022, alors qu'on ne compte que 13 800 agents pour plus de deux millions d'expatriés.

nous notons la dégradation de la qualité des services publics au détriment des Français établis hors de France. Les dernières échéances électorales l'ont d'ailleurs parfaitement illustré, avec de longues files d'attente dans certains bureaux de vote,

on estime que le cumul des congés abandonnés et des heures écrêtées non récupérables et non rémunérées atteint 70 équivalents temps plein.

seulement des agents du ministère à l'étranger sont des fonctionnaires titulaires, pour un tiers de contractuels et un tiers de recrutés locaux.

Pire, les AESH, en cas de changements de département ou d'établissement perdent, faute de statut et de continuité du contrat, le bénéfice de leur ancienneté une généralisation des temps partiels, qui empêche la très grande majorité des AESH de bénéficier du dispositif Sauvadet. À ce titre, et malgré les discours rassurants du ministre de l'éducation nationale et de nombre de nos collègues, la généralisation des accompagnements mutualisés ainsi que des pôles inclusifs d'accompagnement locaux n'améliorent en rien la situation des AESH. Les décisions prises par plusieurs académies ces dernières semaines tendent à confirmer ce que notre groupe avait pressenti : ces mesures de rationalisation constituent un moyen pour les académies de compresser les effectifs et de les réduire drastiquement. Il faut par ailleurs relever que dans les faits, et faute de statut général protecteur, les AESH travaillent à temps complet en participant pleinement à la vie des établissements et en s'autoformant. une concurrence naissante puisque le développement du service civique a conduit certaines académies et établissements à renoncer au recrutement d'AESH et

l'exemple du ministère de la culture. Environ 12 000 des 25 000 agents de la rue de Valois ne sont pas titulaires ; 35 % sont sous contrat à durée déterminée. Cela fait du ministère cher à André Malraux l'un des plus précaires de la fonction publique d'État. Pire,

On en arrive donc à des situations que je n'hésite pas à qualifier de parfaitement stupides. Ainsi, sur certains projets pluriannuels de rénovation ou de restauration, par exemple,

Les recrutements seront prononcés à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics dont les modalités, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'emploi à pourvoir et de la durée du contrat, seront fixées par décret en Conseil d'État. Il n'est donc nul besoin d'imposer de nouvelles procédures, les employeurs devant garder toute latitude en la matière. Il apparaît pour le moins paradoxal de vouloir durcir l'encadrement des conditions de recrutement des agents contractuels au moment où le Gouvernement entend justement leur ouvrir largement l'accès à la fonction publique. Pour tous ces motifs, il convient de supprimer la mesure envisagée. La parole

Dans sa rédaction adoptée par la commission, l'article 6 du projet de loi a pour seul objet d'imposer la règle suivant laquelle, dans la fonction publique d'État, nul ne peut être recruté sur un emploi contractuel dont la création ou la vacance n'a pas été préalablement publiée. Cette règle est déjà satisfaite, dans les deux autres versants,

l'intention de nos collègues est satisfaite, puisque la commission des lois a entièrement réécrit l'article 6 pour supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État censé définir la procédure de recrutement d'agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique et ne maintenir que l'obligation, pour

pour des raisons assez différentes de celles évoquées par Mme la rapporteur, je demande le retrait des amendements n 296 rectifié et 500, considérant qu'il y a un intérêt, notamment pour garantir le principe d'égal accès à l'emploi public, à ce que des dispositions soient prévues pour encadrer le recrutement des contractuels.

l'élargissement des conditions de recours aux agents contractuels dans les trois fonctions publiques doit être accompagné de cette garantie de l'égal accès à l'emploi public pour tous les agents, et donc d'une procédure qui, à défaut d'encadrer et de

j'ai indiqué hier dans la discussion générale que les conditions de travail sur ce texte avaient été particulièrement mauvaises. Je précise, puisque visiblement l'expression de mon agacement a manqué sa cible, que je ne mettais pas en cause le président Bas ou les rapporteurs, dont j'admire le travail dans ces conditions particulièrement difficiles.

secrétaire d'État. Comme je l'ai indiqué précédemment en réponse aux amendements de suppression, le Gouvernement avait prévu dans le texte initial qu'un décret puisse définir les procédures de recrutement des agents contractuels. peut apparaître comme une mesure d'encadrement, et votre commission l'a considérée comme superfétatoire et trop rigide. Je tiens pourtant à souligner l'objectif que nous poursuivons et les raisons qui nous ont conduits à intégrer une telle disposition au texte.

nous avons pris un certain nombre de dispositions réglementaires, parmi lesquelles le décret du 28 décembre 2018, qui met en place un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique, avec une obligation de publicité des offres d'emplois vacants, qu'il s'agisse de postes de titulaires ou de contrats de plus d'un an. Par ce même décret, nous avons établi

J'ai entendu un certain nombre d'interrogations et j'ai pris connaissance des travaux de votre commission sur le sujet. Les employeurs territoriaux, notamment, peuvent craindre que ces procédures ne soient trop rigides. Cela me donne l'occasion de préciser ce que nous envisageons d'intégrer dans le décret en matière d'encadrement de ces procédures de sélection.

la possibilité d'avoir des jurys organisés de manière parfois un peu déconcentrée- Mme la rapporteur connaît parfaitement ce système - : il peut y avoir un jury unique, mais avec des sections différentes lorsque les candidats sont extrêmement nombreux.

élément peut être de nature à rassurer les membres de votre commission et, à travers eux, les employeurs territoriaux -que les procédures de recrutement de contractuels doivent être adaptées à la taille de la collectivité ou de l'établissement qui recrute. Il serait évidemment impensable de prévoir les mêmes procédures de recrutement

que le Conseil constitutionnel, à l'occasion soit d'un examen du projet de loi, soit d'une question prioritaire de constitutionnalité, puisse être puisse être convaincu que ce principe constitutionnel d'égalité devant l'emploi public est respecté, quand bien même nous ouvrons largement les possibilités de recours aux contrats. C'est la raison pour laquelle je sollicite le rétablissement de ces dispositions et, donc, la possibilité de prendre un décret pour

d'égal accès aux emplois publics s'applique au recrutement d'agents contractuels tout autant que de fonctionnaires, il appartient selon nous aux autorités locales de définir la procédure appropriée de recrutement de leurs agents contractuels pour garantir l'effectivité de ce principe, en tenant compte des moyens dont elles disposent, du niveau hiérarchique des emplois concernés, de la nature des fonctions et de la durée du contrat. que l'élargissement du recours aux contrats prévus dans le projet de loi, qui est beaucoup plus modéré dans la fonction publique territoriale que dans la fonction publique de l'État, ne justifie pas que les procédures soient alourdies. Jusqu'à présent, les employeurs territoriaux ont bien su recruter leurs contractuels.

Par analogie, on pourrait considérer que les emplois de direction des collectivités locales sont également à la discrétion de l'autorité politique,

Actuellement, les recrutements contractuels sont possibles dans les communes de plus de 80 000 habitants. Votre texte abaisse ce seuil à 40 000 habitants, ce qui ne change pas la face du monde. S'agissant

la préoccupation de l'égal accès aux emplois publics existe pour l'autorité de nomination, mais on n'est pas obligé de mettre en concurrence des candidats

celui-là même qui est actuellement respecté dans les communes de plus de 80 000 habitants -pour les communes dont le nombre d'habitants est compris entre 40 000 et 80 000.

des recrutements contractuels, qui ne justifie pas de mon point de vue, en contrepartie, qu'un décret vienne limiter dans un nouveau domaine la liberté d'action

les exécutifs locaux disposent d'un pouvoir réglementaire et que l'on pourrait leur faire confiance. D'ailleurs, le contrôle de légalité existe, et s'il leur arrivait de violer un principe aussi fondamental de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que l'égal accès aux emplois publics, le juge administratif ne manquerait pas de les sanctionner et d'annuler les recrutements qui seraient intervenus en violation de ce principe fondamental de la Constitution ! Faisons, s'il vous plaît, confiance aux élus locaux- le Gouvernement s'engage à le faire dorénavant après avoir, il est vrai,

200 agents. Nous respections les règles et il n'y a jamais eu de problème ! Pour les contractuels, en particulier, la règle était parfaitement respectée.

à la manière dont nous traitons en général la question du pouvoir réglementaire des élus locaux. Trop souvent, une compétence donnée aux élus locaux fait l'objet d'un tel encadrement par le pouvoir central et d'une telle défiance

vise à mettre en conformité notre droit avec nos exigences constitutionnelles, dès lors que, d'une part, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame l'égal accès des citoyens aux emplois publics, « sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents d'autre part, l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et aux emplois publics. L'étude d'impact prévoit par ailleurs que, « en l'état du droit, ce n'est qu'en raison de leur caractère dérogatoire que les recrutements d'agents contractuels ne sont soumis au respect de ce principe qu'en tant qu'il requiert la mise en oeuvre d'une procédure de recrutement sous peine d'être entachée d'illégalité Cela suggère donc que l'état du droit pourrait évoluer et qu'aucun principe supralégislatif ne s'oppose à une telle évolution, hormis la volonté du législateur lui-même de prévoir des régimes dérogatoires. Le groupe du RDSE étant très attaché à l'idée de mérite et aux vertus du concours permettant justement une sélection à ce titre, nous ne sommes pas favorables à ce que la notion de mérite disparaisse du fait de la généralisation de recrutements contractuels opaques. Nous considérons au contraire que ces recrutements devraient permettre de retenir des candidats aussi méritants que les candidats aux concours, mais aux qualités ne pouvant être révélées par ce type de recrutement, afin de pallier certains biais culturels.

La rédaction de la commission est déjà très large. Nous avons pourtant volontairement laissé de côté les recrutements de contractuels visant à assurer le remplacement momentané d'un agent occupant un emploi permanent certains emplois qui obéissent à des règles très spécifiques, comme ceux des ouvriers de l'État ou encore des professeurs invités dans les universités, pour lesquels il n'y aurait pas grand sens à imposer une publication préalable ; ou encore les emplois des autorités publiques et administratives indépendantes, qui gèrent leur personnel de manière autonome,

La rédaction de la commission, même si elle ne satisfait pas totalement le Gouvernement, nous paraît suffisamment large dans sa cible. L'objectif que nous poursuivons permettra, je crois, de répondre à votre attente.

Il s'agit de préciser au niveau législatif les modalités de recrutement des agents contractuels afin de garantir effectivement le principe d'égal accès aux emplois publics. Malgré les fondements juridiques de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 34 de la Constitution et la jurisprudence vigilante de Conseil constitutionnel, la loi est restée jusqu'à présent relativement laconique quant aux exigences s'appliquant aux procédures de recrutement d'agents publics contractuels. Les lois de 1984 et 1986 relatives aux trois fonctions publiques prévoient uniquement que les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel les vacances de tous les emplois, hors emplois réservés. Depuis la loi Sauvadet, les exigences ont été renforcées pour les emplois de la fonction publique territoriale, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération devant être précisés dans les offres publiées. Compte tenu de la volonté d'accroître le recours aux agents contractuels, il importe de rendre le principe d'égal accès plus effectif, en prévoyant davantage de garanties dans la loi pour les trois versants de la fonction publique. Au nom de quel principe les garanties prévues en matière de fonction publique de l'État seraient-elles moins précises que celles prévues en matière de fonction publique territoriale ? Le présent amendement vise donc à introduire dans la loi des dispositions applicables aux trois versants, destinées à garantir l'organisation effective d'une procédure de recrutement et à éviter le fléchage de postes vers des candidats en réalité présélectionnés. Quel

pour pourvoir des emplois permanents de l'État et de ses établissements publics est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. L'auteur de l'amendement, Mme Delattre, propose d'ajouter que cette publication doit s'effectuer « en ligne